parole est à M. Antoine Lefèvre. Cet amendement vise à étendre aux transports publics de voyageurs du quotidien, c'est-à-dire aux transports publics urbains et régionaux, y compris les transports scolaires et les transports spécialisés pour les personnes en situation de handicap, le taux appliqué aux produits de première nécessité. En effet, le rôle essentiel des transports publics de voyageurs pour favoriser la mobilité de tous et lutter contre les exclusions n'est plus à démontrer. Il est donc primordial que les transports publics soient désormais considérés comme un service de première nécessité. Quel est l'avis de la commission ?

2012. Le 1 janvier 2012, le taux de TVA applicable à ces parcs est passé à 7 %, avant d'être porté à 10 % au 1 janvier 2014, ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement trois Il s'agit d'un amendement de cohérence et d'égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d'activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des spectacles vivants. Ainsi, les cirques

Une enquête indique que le retour au taux réduit de 5,5 % est un enjeu majeur de croissance et de création d'emplois, si ce n'est de pérennité de l'activité de ce secteur.

dans la nature, mais également des moteurs de recherche et de conservation des espèces animales. Aussi, compte tenu, d'abord, de la possibilité de gager sur les droits sur les alcools le faible manque à gagner pour l'État qui résulterait de l'assujettissement des parcs zoologiques au taux réduit de 5,5 %, et, ensuite, de l'important bénéfice pour l'emploi, le développement et l'investissement

Cette augmentation avait été décidée pour financer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui n'a pas porté les fruits escomptés en matière d'emploi. En revanche, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement sentir dans les budgets des collectivités territoriales et, en conséquence, sur les impôts locaux des habitants. L'application du taux de 10 % a en effet fait doubler le poids de la TVA en deux ans, ce qui pèse directement sur le pouvoir d'achat des Français, à hauteur de 150 millions

maintient les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle dans le périmètre des variables d'ajustement et accentue leur diminution. L'article 15 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, codifié à l'article 1648 A du code général des impôts, complété par le décret du 17 octobre 1988 relatif aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, a institué les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Ces fonds ont pour objet de répartir dans chaque département les produits de la taxe professionnelle des grands établissements industriels entre la commune d'implantation, les communes proches et les communes défavorisées du département. Le conseil départemental octroie les fonds aux communes défavorisées selon les critères qu'il a fixés.

monsieur Dantec,

et souligne le travail extrêmement important effectué au sein de la commission des finances sous la houlette du rapporteur général. Nous tenons à rappeler la nécessité d'agir urgemment sur le sujet. En effet, le commerce en ligne est en train de se développer à très grande vitesse et les risques de perte de recettes pour l'État sont très importants.

il serait bon que l'on puisse adopter cet amendement à l'unanimité.

fait de la décision rendue le 19 mai 2017 par le Conseil constitutionnel, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit de revoir les modalités de calcul et de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. la règle de calcul du taux effectif en fonction du chiffre d'affaires des sociétés membres d'un groupe intégré serait ainsi étendue aux sociétés qui ne sont pas membres d'un groupe, mais qui remplissent les conditions liées à la détention pour en faire partie. Seraient ainsi concernés tous les groupes dans lesquels les conditions de détention, directe ou indirecte, à 95 % du capital seraient remplies. Comme dans le régime antérieur, la consolidation ne serait pas pratiquée lorsque la somme du chiffre d'affaires est inférieure à 7,63 millions d'euros. Or, il n'y a pas de fondement à retenir un calcul du chiffre d'affaires consolidé uniquement parce que des entreprises ont un lien capitalistique et constituent seulement un groupe économique. Les sociétés restent indépendantes. Cette extension du périmètre de l'entreprise mère aura des conséquences pour un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont plusieurs sociétés. En outre, l'article 7 du projet de loi de finances prévoit de porter le coefficient de pondération des immobilisations industrielles de 5 à 21, sans en expliciter le motif.

l'activité et l'égalité des chances économiques, les entreprises réalisant un investissement productif éligible ont bénéficié jusqu'au 14 avril 2017 d'un avantage fiscal leur permettant de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient de cet investissement. Ce suramortissement s'ajoutait à l'amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun. Contrairement à une mesure d'accélération du rythme de déduction de l'amortissement, il ne s'agissait pas seulement de procurer un gain de trésorerie à l'entreprise, l'économie d'impôt réalisée étant définitive. Ce dispositif a rencontré un franc succès et a permis de relancer l'investissement dans de nombreux secteurs productifs, investissement dont notre industrie a cruellement besoin étant donné son retard dans ce domaine, notamment par comparaison à sa concurrente allemande. Toutefois, Toutefois, la loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016 dispose que ces investissements devaient être réalisés ou engagés avant le 15 avril 2017. Nombre d'entreprises qui souhaitent aujourd'hui investir hésitent à aller au bout de leur démarche du fait de la disparition de cet avantage fiscal. Cet amendement prévoit de rouvrir le dispositif pour un an en ciblant spécifiquement les investissements susceptibles de favoriser la mécanisation, la robotisation et la numérisation, afin de soutenir la nécessaire transition de l'industrie française

C'est un excellent levier d'aide à l'investissement pour les entreprises industrielles, qui se tournent vers l'industrie du futur et concourent ainsi à la réindustrialisation très attendue de nos territoires.

de vote. Monsieur le ministre, nous avons en effet un désaccord structurel sur la manière de concevoir l'avenir de l'industrie française. On peut avoir tous les débats du monde sur l'impact de la baisse du coût du travail sur la compétitivité globale de l'économie.

« était sans doute nécessaire d'aider les entreprises à reconstituer leurs marges avec le CICE. La réduction du taux de l'impôt sur les sociétés va permettre d'aller plus loin dans cette direction. »

soit 29,1 millions de tonnes équivalent pétrole. Le discours du Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès le 3 juillet 2017 et la déclaration de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée nationale le 4 juillet 2017 ont clairement réaffirmé les ambitions de la France en matière de production d'énergies renouvelables, qui doivent représenter 23 % de la consommation brute d'énergie en 2020. Les nécessaires investissements sur les territoires en matière de production d'énergies renouvelables doivent donc être accélérés par la remise en route de ce dispositif fiscal, qui a fait ses preuves. Cette disposition jouerait également un rôle de catalyseur pour renforcer l'indépendance énergétique de la France à l'égard des sources d'énergie non renouvelables.

par un décret du 14 septembre 2007. Ce titre est délivré par le préfet du département pour une durée de quatre ans sur la base d'un audit de conformité réalisé par des organismes certificateurs agréés, indépendants et dont la compétence en matière de restauration traditionnelle est incontestée. ouvre droit à un crédit d'impôt de 50 % des dépenses de modernisation engagées sur une durée maximale de trois ans et pour un montant maximal de 30 000 euros. Le crédit d'impôt peut ainsi atteindre 15 000 euros.

du titre de maître-restaurateur demeure en phase de développement. Les titulaires demeurent insuffisamment nombreux au regard du nombre de professionnels remplissant les conditions requises. Afin de continuer à soutenir le développement du dispositif, il est nécessaire de maintenir le crédit d'impôt, qui revêt, pour les professionnels et leurs représentants, un aspect incitatif déterminant. Sa fin entraînerait un risque d'arrêt brutal du développement du titre de maître-restaurateur et condamnerait ainsi la politique suivie en faveur du développement de la qualité dans les établissements de restauration traditionnelle. Il est donc proposé de proroger ce dispositif, qui doit prendre fin le 31 décembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2020. Quel Quel est l'avis de la commission ?

la politique écologique recoure abusivement à la fiscalité. Depuis toujours, nous combattons ce que nous appelons la fiscalité punitive. Or c'est malheureusement

Cet amendement vise à exonérer le carburant biométhane de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, pour mettre en cohérence l'ensemble de la fiscalité sur le biométhane, quel qu'en soit l'usage.

porte sur le carburant ED95, qui est destiné à des flottes captives de bus ou de poids lourds ne pouvant fonctionner qu'avec ce carburant composé à 95 % de bioéthanol et à 5 % d'un additif dilué dans de l'eau. L'augmentation de la TICPE le carburant ED95 va désavantager celui-ci par rapport au gazole, qui bénéficie d'un plafonnement de TICPE pour les transporteurs routiers.

pour faire un effort déjà significatif pour 2018, mais mettons ensemble nos capacités à travailler pour associer

elles soient exonérées des efforts ou de l'envie de participer parce qu'elles ont moins de 20 000 habitants. Relevons ensemble ce défi. Nous y sommes prêts, monsieur le ministre

Cet amendement vise, d'une part, à introduire le B100 dans la nomenclature de l'article 265 du code des douanes en créant un nouvel indice 57, et, d'autre part, à lui appliquer un taux de TICPE limité à sa seule composante correspondant à la contribution climat-énergie, sur le même modèle que celui qui a été prévu pour l'ED95. Une telle mesure contribuera également à réaliser, d'ici à 2020, les objectifs européens de 10 % d'utilisation d'énergies renouvelables dans le secteur des transports et de 20 % d'énergies renouvelables dans le bouquet énergétique total, conformément à la directive 2009-28-EC. J'ai bien entendu les demandes et les propositions du rapporteur général sur ce point. Toutefois, j'aurais souhaité une trajectoire beaucoup plus longue. Ce que je voudrais souligner- cela a été dit pertinemment tout à l'heure par notre collègue Cuypers -, c'est que cette filière est le fruit d'un engagement de l'ensemble de la profession agricole, de ceux qui ont créé cette filière oléoprotagineuse qui nous est enviée par beaucoup de pays membres de l'Union Or les entreprises, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, mais surtout dans celui-là, ont besoin de lisibilité. La lisibilité, c'est la stabilité et la durabilité législatives. voudrais vous rappeler, au travers des externalités positives, que c'est un subtil équilibre entre du biocarburant, de la protéine végétale et un secteur émergent extrêmement porteur, celui de la chimie verte.

dont la consommation en énergie est souvent contrainte. En outre, comme l'Observatoire français des conjonctures économiques le rappelle, la localisation des ménages est une autre source d'inégalité face à la taxe carbone, en raison de l'usage plus important de l'automobile en milieu rural ou dans les communes de moins de 30 000 habitants.